La séance est reprise. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis heureux de saluer en votre nom, la présence dans la tribune d’honneur, du président du Sénat de la République démocratique du Congo, M. Sama Lukonde, et d’une délégation de sénatrices et de sénateurs, dont le président de la commission des relations extérieures et celui de la commission de la défense. Ils sont accompagnés par nos collègues Guillaume Chevrollier, président du groupe d’amitié France Afrique centrale, et Francis Szpiner, président délégué pour la République démocratique du Congo. Nous venons de l’évoquer avec le président du Sénat de la République démocratique du Congo : alors que celle ci connaît une situation humanitaire dramatique, du fait, en particulier, des tentatives de déstabilisation orchestrées dans l’est du pays par le Mouvement du 23 mars (M23) et le Rwanda, le Sénat assure le peuple congolais de sa solidarité et de son attachement indéfectible à son intégrité territoriale

2773 condamnant les offensives du M23 et appelant au cessez le feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous tenons à le rappeler avec force : la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne sont pas négociables. Il y va de la stabilité du continent africain tout entier, nous venons de l’évoquer et de le partager.

Mes chers collègues, en votre nom à tous, je souhaite à nos collègues de la République démocratique du Congo des échanges riches et féconds, en les assurant de l’amitié et de la confiance du Sénat de la République française.

chers collègues, avant de passer à notre ordre du jour, je voulais vous faire part d’un incident grave qui s’est produit lors de la séance du mardi 18 février après midi, au cours des débats sur la proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Alors que le président Patrick Kanner avait la parole pour explication de vote sur les amendements portant suppression de l’article 1 de la proposition de loi, notre collègue Stéphane Ravier est intervenu en employant notamment le mot de « collabo » à son encontre. Laurent Burgoa a pris la parole en séance pour confirmer l’emploi de ce terme, comme l’atteste le compte rendu des débats. Ces propos, qui ont été entendus par d’autres de nos collègues, sont constitutifs d’une injure et sont donc passibles de la censure aux termes de l’article 94 de notre règlement. Par une lettre en date du 19 février 2025, le président Patrick Kanner m’a donc demandé de prononcer cette sanction contre Stéphane Ravier, qui emporte, de droit, la privation, pendant un mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction. Jamais la censure n’a été prononcée contre un sénateur sous la V République. Le bureau du Sénat s’est réuni le jeudi 20 mars afin d’examiner la situation de Stéphane Ravier. Le caractère inacceptable du propos tenu par notre collègue a fait l’objet d’un consensus unanime. Dans le cadre de la procédure, Stéphane Ravier a toutefois, par écrit, reconnu les faits et a présenté ses excuses au Président Kanner. Au regard de ces éléments, et après consultation du bureau, j’ai donc décidé de ne pas proposer au Sénat de prononcer la censure, mais de procéder à un rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal. J’adresse donc ici un rappel à l’ordre avec inscription au procès verbal à Stéphane Ravier pour son attitude à l’égard du président Patrick Kanner lors des débats sur la proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport. Mes chers collègues, je me fais ici l’interprète du bureau du Sénat, là encore unanime, pour appeler solennellement chacune et chacun d’entre vous, dans tous les groupes, au respect mutuel. Des débats difficiles nous attendent ces prochains mois et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, basculer dans les injures et les outrages. Méfions nous des mots à charge polémique

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement, présentée par M. Khalifé Khalifé

nous examinons aujourd’hui la proposition de loi visant à convertir les centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique

mes chers collègues, de saluer les nombreux salariés de cette centrale, ainsi que les élus du bassin de Saint Avold qui, accompagnés du président du conseil départemental de la Moselle, M. Patrick Weiten, ont fait le déplacement au Sénat en cette journée cruciale. insiste, car le sujet que nous traitons aujourd’hui dépasse la simple question énergétique : il s’agit d’emploi, de justice sociale et de responsabilité envers des territoires comme la Moselle qui ont fait, deux siècles durant, la force industrielle de la La centrale Émile Huchet est un symbole de cette histoire. Sa dénomination est un hommage à celui qui dirigea la compagnie des houillères après le retour de ces territoires annexés à la France. Construite au pied des mines à la sortie de la guerre et dans l’esprit du programme du Conseil national de la Résistance (CNR), cette centrale, qui fut l’une des plus importantes d’Europe, a joué un rôle clé dans notre approvisionnement énergétique. Aujourd’hui, elle est l’un des témoins de cette grande aventure industrielle.

qui, encore récemment, n’ont pas hésité à rallumer la flamme pour que nous ayons de l’électricité alors que la guerre et la crise frappaient de nouveau l’Europe.

: il nous faut stabiliser les emplois et sécuriser les dizaines de millions d’euros d’investissement nécessaires à cette conversion demandée en 2023 par le Président de la République. Cette Cette promesse, nous devons désormais la réaliser : tourner la page du charbon sans reproduire les erreurs et sans tolérer les stigmates, encore visibles, laissés par les politiques publiques mises en œuvre lors de la fermeture des mines de charbon et des aciéries.

Nous devons faire de l’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon un exemple en termes de transition énergétique, sociale, environnementale et industrielle. Cette proposition de loi, que j’ai déposée avec l’ensemble de mes collègues de Moselle, au delà de toute appartenance politique, également cosignée par les sénateurs lorrains et par plusieurs dizaines d’autres sénateurs, que je remercie chaleureusement. Solution pragmatique et équilibrée, elle permet une conversion rapide des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs, comme le gaz et le biogaz, sans peser sur les finances publiques. Elle garantit le maintien des emplois, tout en réduisant les émissions de CO2 d’un facteur 2 à 3. En un mot, elle concilie l’exigence écologique avec la nécessité économique et sociale. Résultat d’un consensus construit entre les collectivités, les parlementaires, le Gouvernement, l’exploitant et les salariés du site, elle permettra de poursuivre la sécurisation du système électrique lors des pointes de consommation, en particulier en cette période

environ un an. La conversion permettra de maintenir une centrale d’une capacité de 600 mégawatts et sécurisera le système électrique national. Cette solution technologique

les modifications du texte initial, plus spécialement celles qui concernent le périmètre, ne nous ont guère rassurés quant à la viabilité et à la pérennité, même à moyen terme, de l’investissement humain et financier prévu.

par une bonne intention, à savoir sécuriser le dispositif, les modifications proposées risquaient à nos yeux de transformer un processus de conversion efficace en un labyrinthe qui aurait condamné cette centrale à la fermeture. Notre proposition de loi comportait initialement deux articles. Le premier vise à reconnaître que l’installation, une fois convertie, est une nouvelle installation de production, permettra de candidater au nouveau mécanisme de capacité. Le deuxième article permet d’octroyer une autorisation de production à la centrale à charbon une fois convertie, si elle est lauréate du nouveau mécanisme de capacité. Je tiens à vous préciser, mes chers collègues, que cette proposition de loi est en adéquation avec la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) actuellement soumise à la consultation, et qui fait de Saint Avold un site pilote en la matière.

Lors de l’une de mes visites dans cette centrale, j’ai été profondément marqué par cette phrase d’un salarié : « Une transition bien pensée est celle qui ouvre une porte sans en fermer une autre brutalement. Cela résume parfaitement l’enjeu de notre débat, mes chers collègues : nous voulons sortir du charbon, mais nous devons le faire en garantissant un avenir aux salariés et aux territoires concernés. Cette proposition de loi sera donc un réel test de notre volonté politique de respecter les engagements pris devant nos concitoyens et de leur offrir un avenir stable. Aujourd’hui, nous avons la possibilité de faire un choix historique. En adoptant cette proposition de loi, nous enverrons un message clair : oui, la transition écologique peut être socialement juste et économiquement viable. Mes chers collègues, nous avons une énorme responsabilité et devons être à la hauteur des enjeux, qui sont majeurs. Ne répétons pas les erreurs du passé : toute la France se souvient encore de la fermeture du site de Florange, en Moselle, et de ses conséquences humaines et politiques… Comme vous, je sais combien la Haute Assemblée est attachée à la défense de nos territoires. En votant cette proposition de loi et nos amendements, vous aurez l’occasion de réaffirmer votre engagement et de confirmer l’une des missions du Sénat

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que nous soyons réunis aujourd’hui pour examiner un texte transpartisan

Je rappelle que ce projet concerne 500 emplois, directs ou indirects, dans un département, la Moselle, durement éprouvé par la fermeture des mines de charbon.

Sur cette base, un décret du 5 février 2022 et une ordonnance du 29 juillet 2020 ont été pris. Compte tenu de la crise des prix des énergies entre 2022 et 2023,

Le Havre et Gardanne, ont été fermées en 2021, tandis que deux autres, Cordemais et Saint Avold, étaient maintenues. Dans le cadre de la révision de notre programmation énergétique, qui est toujours en cours, le Gouvernement envisage un objectif de sortie ou de conversion des deux dernières centrales à charbon d’ici à 2027,

prévoit de « fixer les conditions de fermeture ou de conversion […] des dernières centrales à charbon, qui doivent être effectives au plus tard en 2027 Ensuite, le projet de programmation pluriannuelle de l’énergie, soumis à consultation publique, vise, d’une part, à « organiser et accompagner la fin de la production d’électricité à partir de charbon » et, d’autre part, à « accompagner le lancement d’études ou de sites pilotes […] pour la conversion de centrale thermique Dans cette perspective, une centrale, en l’occurrence celle de Saint Avold, pourrait être convertie. La proposition de loi vise à favoriser la conversion des centrales à charbon dans le cadre du mécanisme de capacité. Réformé par la loi de finances pour 2025, ce mécanisme consiste en un dispositif de rémunération, par Réseau de transport d’électricité (RTE), des exploitants de capacités de production en contrepartie de leur engagement de disponibilité. Pour le financer, une taxe sur les fournisseurs et les consommateurs d’électricité est affectée à RTE. Comme le précédent dispositif, le nouveau mécanisme de capacité doit être notifié par la France à la Commission européenne au titre des aides d’État.

De son côté, l’article 2 vise à regrouper les autorisations des centrales à charbon faisant l’objet d’une conversion dans le cadre du mécanisme de capacité. À cette fin, il dispose que la sélection par ce mécanisme tient lieu de l’autorisation d’exploiter prévue par le code de l’énergie. En dépit d’un calendrier contraint, j’ai organisé six auditions et reçu six contributions, recueillant ainsi les points de vue de l’ensemble des parties prenantes. J’en retiens que ce texte est accueilli favorablement.

La direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), RTE et la Commission de régulation de l’énergie (CRE) m’ont aidé dans cette tâche. Nous devons être très vigilants quant à la robustesse du texte, car la précédente autorisation des centrales à charbon, mal calibrée, a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en 2022. Il ne faut absolument pas que ce scénario se reproduise, car cela remettrait durablement en cause les projets d’investissements prévus. Le texte adopté en commission laisse inchangé le périmètre initial de la proposition de loi, qui concerne les énergies fossiles. Dans ce contexte, il pourrait aussi servir d’appui à un projet de conversion vers les huiles végétales hydrotraitées, expérimenté à la centrale de Vaires sur Marne. Si nous avons laissé ce périmètre tel quel, c’est parce que le règlement sur le marché intérieur de l’électricité de 2019, tel qu’il a été révisé en 2024, applique un même seuil d’émissions à toutes les énergies fossiles. le texte adopté en commission aucune nouvelle contrainte et aucun nouveau délai. Nous avons introduit une référence à la loi de finances pour 2025, car le mécanisme de capacité auquel la proposition de loi raccroche les centrales à charbon doit, selon ladite loi, entrer en vigueur après notification auprès de la Commission européenne au titre des aides d’État. Le Gouvernement nous a rappelé que les négociations étaient déjà en cours, la notification du dispositif devant intervenir en 2025 et son application d’ici à 2026. Tel est le droit existant. Nous avons aussi introduit une référence au code de l’environnement, car le regroupement des procédures proposé, entre l’autorisation d’exploiter prévue par le code de l’énergie et la sélection du mécanisme de capacité, n’a pas vocation à supprimer les exigences environnementales.

précisé que le texte concernait les seules centrales existantes et non les nouvelles. L’objectif de la proposition de loi est de faciliter la conversion des installations existantes et non de déroger à l’article 8 du décret du 21 avril 2020 relatif à l’actuelle PPE, qui prohibe les nouvelles installations. Une telle précision présente un double intérêt : sur le plan économique, elle évite que les projets de reconversion soient évincés au profit de nouveaux projets et protège Saint Avold ; sur le plan environnemental, elle constitue un garde fou utile, les nouvelles capacités de production d’électricité devant être nucléaires et renouvelables. D’autre part, avec mon appui, nous avons ajouté une disposition demandant au groupe EDF de préciser le devenir de la centrale à charbon de Cordemais. Au nom de notre commission, je vous invite donc à adopter cette proposition de loi. Soyez assurés de ma détermination sans faille à la faire aboutir dans le cadre de la navette parlementaire

trouve son origine dans l’urgence de sauvegarder les emplois de la centrale thermique à charbon de Saint Avold, en Moselle. En permettant la conversion de cette centrale à charbon vers une source d’énergie moins polluante, cette proposition de loi représente un petit pas pour l’environnement et un grand pas pour l’emploi. l’emploi. Très attendue par les élus et les habitants du département, elle me tient particulièrement à cœur. Je tiens ici à saluer la présence des salariés, des sous traitants,

Avec mes collègues sénateurs de Moselle, nous avons pris l’initiative de présenter ce texte pour défendre la vitalité économique de notre département. Alertée il y a quelques mois sur l’urgence de cette reconversion, j’avais interpellé le Gouvernement, qui m’avait encouragée à légiférer sur Le choix d’un dépôt collectif traduit notre engagement commun, l’ordre de signature des auteurs ayant été déterminé par âge décroissant. d’un texte de circonstance, porteur de beaucoup d’espoirs pour les 150 salariés de cette centrale, les 150 sous traitants et les 500 emplois directs et indirects du territoire. Depuis l’annonce en 2019 de la fermeture progressive des centrales à charbon, ces travailleurs vivent dans une incertitude permanente. Cette situation est inacceptable. Ils ont tout connu : une fermeture en février 2022, votée dans cet hémicycle ; une réouverture quelques mois plus tard, votée en urgence une fois ; l’échec d’un projet de conversion à la biomasse ; enfin, un projet de conversion au gaz et au biogaz. Il est, dans ce contexte, de notre responsabilité d’envoyer un signal clair à ces salariés, trop souvent soumis aux aléas des décisions politiques. La fermeture des centrales thermiques à charbon est une nécessité. Aujourd’hui, 95 % de la production d’électricité en France est bas carbone grâce à notre parc nucléaire et au développement des énergies renouvelables. Le charbon ne représente plus qu’une part infime

après sa fermeture. Puis, en septembre 2023, le Président de la République a annoncé la conversion des deux dernières centrales à charbon d’ici à 2027. Cet engagement, nous le devons aux salariés. L’exploitant a proposé une conversion au gaz naturel et au biogaz, soutenue par le ministre de l’économie, le 12 février dernier. Nous en convenons, le gaz naturel reste une énergie fossile et n’est pas la solution optimale ; il constitue malgré tout un progrès, étant deux fois moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon. De surcroît, la centrale n’a pas vocation à fonctionner en continu. Elle interviendra en période de pointe, garantissant ainsi la stabilité du réseau électrique et une sécurité d’approvisionnement électrique en hiver, soit l’équivalent de quatre semaines de production par an. Enfin, nous devons toujours concilier environnement et justice sociale. Ce projet est une solution de compromis qui assure la préservation des emplois tout en réduisant l’empreinte carbone de la production électrique.

en accédant au nouveau mécanisme de capacité. La commission d’aménagement du territoire et du développement durable a émis un avis favorable sur la proposition de loi

madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui nous réunit aujourd’hui est porteuse d’espoir et de solutions. Notre pays doit une partie de son histoire au charbon. Au moment de sortir ce combustible de notre production d’électricité, je souhaite rappeler qu’entre 1230 et 2004, le charbon a fait vivre des bassins entiers de population. Le pacte charbonnier, négocié en 1994, avait permis un arrêt progressif de l’extraction houillère. La dernière mine profonde à fermer était celle de La Houve, en Moselle, en 2004. L’accompagnement des territoires et des anciens mineurs avait été la clé de voûte de ce pacte. Accompagner

Avec elle, c’est l’avenir de nombreuses familles et de tout un territoire qui est en jeu. Si ce texte est porteur d’espoir, c’est parce qu’il est porteur de solutions. Il s’agit de convertir cette centrale à charbon vers un combustible beaucoup moins émetteur en dioxyde de carbone : le biogaz.

Elle confirme l’attachement du Sénat au dynamisme de nos territoires et témoigne de la culture du dialogue, qui est la marque de fabrique de cette assemblée. Je salue, en particulier, la mobilisation des sénateurs mosellans Khalifé Khalifé, Christine Herzog, Jean Marie Mizzon, Catherine Belrhiti et Michaël Weber, ainsi que l’engagement des élus de Moselle et de la région Grand Est. Le Gouvernement soutient pleinement cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie nationale en faveur de la transition énergétique à l’échelle des territoires. En septembre 2023, le Président de la République avait pris l’engagement de convertir les centrales à charbon françaises afin de réduire nos émissions de dioxyde de carbone et de garantir la sécurité d’approvisionnement électrique de notre pays. la centrale de Saint Avold ont ainsi présenté un projet de conversion de la centrale au biogaz. De nombreux échanges ont eu lieu depuis lors avec mes services afin de préciser les modalités de cette conversion.

Ce texte vise à garantir que les centrales à charbon converties à une autre source d’énergie primaire, moins émettrice, soient éligibles au futur mécanisme de capacité. Parmi les projets concernés, les lauréats seront ceux qui répondent aux besoins de notre pays en matière de sécurité d’approvisionnement électrique.

En l’élargissant à d’autres combustibles fossiles, pour lesquels le coût de conversion serait négligeable, le risque est grand de créer un effet d’aubaine injustifié, qui ferait manquer l’objectif de la proposition de loi : accompagner la défossilisation de notre économie. Cette solution représente une avancée à double titre : elle allège le cadre administratif sans alourdir le budget de l’État. C’est, je crois, assez rare pour être souligné. Naturellement, les projets de conversion demeurent soumis au respect de la réglementation européenne et du code de l’environnement. Pour la centrale de Saint Avold, je sais que les discussions avec les services de l’État sont bien avancées et je puis vous assurer que mes équipes suivent le projet avec beaucoup d’attention. Les bénéfices de cette conversion seront nets et très significatifs. D’abord, pour l’emploi : cette conversion représente un investissement de plusieurs dizaines de millions d’euros de la part de GazelEnergie. C’est une excellente nouvelle pour l’avenir de ce site industriel et pour les 500 personnes, sous traitants compris, dont l’activité est liée à la centrale de Saint Avold. Je salue, à ce titre, les mesures prises par GazelEnergie en faveur des salariés dans cette période délicate de transition, en particulier la prolongation des contrats de travail jusqu’au 31 août 2025, à la demande des organisations syndicales. Les bénéfices sont réels aussi pour notre souveraineté énergétique et pour nos objectifs climatiques. En effet, cette conversion permet de maintenir un avantage qui a son importance, celui de produire de l’électricité dans les périodes de pic de consommation, en complémentarité avec les sources d’énergie renouvelable.

Je garde à l’esprit la situation de cette centrale, dont le projet de conversion à la biomasse n’a pu aboutir en raison de coûts extrêmement élevés. Nous sommes donc pleinement mobilisés, avec EDF, pour assurer le reclassement intégral des salariés, notamment en lien avec l’usine Framatome située à proximité.

démarche transpartisane, de pragmatisme et d’efficacité. Je suis heureux et fier, au nom du Gouvernement, d’apporter mon plein soutien à ce texte porteur d’espoirs et de solutions pour ces hommes et ces femmes engagés dans le grand chantier de la transition énergétique. Bravo ! La parole

à charbon. La transition énergétique demande de l’accompagnement. Il faut une ligne directrice, mais on ne peut bien faire qu’avec les acteurs locaux, les élus et les riverains, afin de créer une dynamique de territoire et, surtout, de l’engagement. Donner les moyens de la transition, c’est à la fois accompagner financièrement et construire une culture du consensus autour de projets et de bénéfices partagés.

On aurait pu imaginer que huit ans suffiraient pour assurer une transition en douceur, mais non : aucune anticipation, aucun accompagnement, aucune stratégie. Disons le clairement, nous payons aujourd’hui l’impréparation et l’absence de vision du Gouvernement sur l’énergie. Il reste deux centrales à charbon en France, à Cordemais et à Saint Avold. Elles représentent environ 1 000 emplois directs et indirects, soit 1 000 salariés qui risquent de se retrouver sur le carreau.

la biomasse, mais sans épuiser nos terres, sans importer d’engrais azotés produits par des énergies fossiles, sans altérer la production alimentaire. Ne répétons pas le fiasco de la centrale Provence 4 de Gardanne : rendement médiocre, étude d’impact bâclée, risque pour les forêts environnantes, annulation de l’autorisation cette centrale, nous importons massivement du bois brésilien : déforester l’Amazonie et le Cerrado pour produire de l’électricité à Gardanne, clairement, cela ne va pas

mais nous devons faire mieux qu’ailleurs. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires appelle le Gouvernement à mettre en place des plans de transition territoriaux avec les entreprises, les salariés et les élus locaux, pour accompagner en douceur le changement, former les salariés, élaborer des calendriers réalistes et des solutions réellement renouvelables. La conversion au gaz est un leurre qui ne pourra durer que quelques années si l’on veut respecter les engagements de l’accord de Paris et sortir de notre dépendance énergétique.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera majoritairement contre ce texte si l’inclusion des centrales au fioul est maintenue dans le dispositif. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons. La parole est à M. Franck

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain,

de donner un contenu juridique à des décisions et à des promesses faites au cours des dernières années, notamment par le Président de la République. Son caractère transpartisan – je salue les sénateurs mosellans qui la soutiennent – nous permettra, je l’espère, de trouver un consensus pour contribuer à l’équilibre du système de production nationale

2035 et 2050 n’a obtenu aucune réponse à cette question. Il y va pourtant du niveau des prix, de leur stabilité et de leur visibilité pour toutes les catégories de consommateurs.

Je pense particulièrement à Cordemais et à Gardanne, qui devraient faire l’objet d’un soutien particulier de la part de l’État. Au risque de me répéter, rien ne nous garantit d’être définitivement à l’abri d’une envolée des marchés de l’électricité similaire à celle qui a été provoquée par l’agression russe contre l’Ukraine en 2022.

il s’agit là d’un véritable déni de démocratie. Comment est il possible que l’énergie, pourtant au cœur de la transition écologique, facteur clé de notre souveraineté nationale future, soit ainsi soustraite à la discussion des représentants de la Nation ?

Les difficultés politiques engendrées par la dissolution de l’Assemblée nationale ne doivent pas servir de prétexte au contournement du Parlement. La parole

monsieur le ministre, mes chers collègues, la raison d’être et le sujet de cette proposition de loi proviennent du fameux cas d’espèce de la centrale à charbon de Saint Avold, dignement défendue, avec énergie, par mon collègue député Alexandre Loubet ainsi que par l’ensemble du mouvement auquel j’appartiens. Saint Avold, c’est tout un symbole des petits calculs politiciens du Président de la République et de la Macronie. En effet, alors que la centrale est fermée en mars 2022, en pleine campagne présidentielle et à quelques jours du premier tour des élections, elle est finalement rouverte à la fin du mois de juin 2022, soit une semaine après le second tour des législatives.

Au Rassemblement national, face au lobbyisme « décroissantiste » des écologistes, qui souhaitent ramener la France à l’âge de pierre, nous avons toujours maintenu le cap : développer le nucléaire, l’énergie la plus décarbonée qui soit, pour nous permette de conserver un maximum de souveraineté.

Nous saluons bien naturellement cette initiative législative transpartisane, même si le Rassemblement national a été bien seul pour défendre Saint Avold. Bien sûr… Toutefois, je tiens à alerter sur l’aberration de la version du texte issu des travaux de la commission, qui menace clairement la faisabilité de la conversion du site et l’avenir des emplois.

Si les sénateurs ne reviennent pas sur ces diverses modifications, ils auront trahi la promesse de favoriser la conversion des centrales à charbon françaises. Dans tous les cas, comme depuis 2022, les salariés de la centrale à charbon de Saint Avold savent pouvoir compter sur le Rassemblement national, au Sénat et à l’Assemblée nationale, pour les défendre.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, des années d’atermoiement et de renoncement, des erreurs parfois guidées par des opportunités politiques, des crises menaçant la sécurité des approvisionnements et mettant en question nos choix passés : tout cela montre

Ne manquons toutefois ni de réalisme ni de vision : seul un cap sur le long terme nous permettra de rendre attractives nos filières, de laisser la porte ouverte aux innovations futures et d’avoir un mix énergétique décarboné, permettant un approvisionnement stable.

auront également des effets sur notre approvisionnement énergétique national. Il y va de notre souveraineté. Le contexte géopolitique l’a montré, nous devons gagner en autonomie.

pour permettre une stabilité du réseau électrique lors des pointes. Par ailleurs, le regroupement des procédures permettant d’établir que la désignation de ces centrales par RTE emporte l’attribution de l’autorisation d’exploiter est une simplification bienvenue. La précision du rapporteur concernant l’autorisation environnementale y participe également. Malgré ces avancées notables, le chemin est encore long. Le vrai défi de demain est technologique, industriel, financier et humain. Nous devons analyser nos échecs et en tirer les enseignements. La consommation croissante d’électricité, le changement climatique et le contexte géopolitique nous obligent à accroître notre production d’énergie décarbonée. Mettons toutes les chances de notre côté. La transformation de notre mix énergétique impose de disposer d’énergies renouvelables intermittentes et d’énergies bas carbone pilotables, puissantes et bien implantées. Toutes ces énergies sont complémentaires pour assurer une production d’énergie continue ainsi qu’un approvisionnement suffisant et régulier, sans affecter durablement notre environnement. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires est toujours investi quand il s’agit de soutenir la souveraineté énergétique de la France.

effets, dite loi Climat et Résilience, l’État a voulu modifier le droit social appliqué aux centrales à charbon. Ici encore, nous avons accompagné ce mouvement sous conditions, en consolidant le droit au reclassement.

Ces projets ne sont pas affectés par les délais d’application du texte, qui doivent être les plus courts possible. La proposition de loi modifie le mécanisme de capacité qui, en application de la dernière loi de finances, fait l’objet de négociations européennes en cours.

en mémoire que la précédente réautorisation des centrales à charbon, mal calibrée, a été partiellement censurée par le Conseil constitutionnel en 2022.

Comme de nombreux collègues, je déplore que le Gouvernement envisage de publier par décret la programmation pluriannuelle de l’énergie, sans passer par la loi de programmation pourtant requise depuis la loi Énergie

du célèbre d’Émile Zola à la chanson de Pierre Bachelet, l’extraction du charbon semble appartenir à une autre époque. Pourtant, force est de constater que le charbon est toujours un sujet d’actualité. Après avoir eu un rôle fondamental dans le développement industriel de la France au XIX siècle, le charbon a été pointé du doigt en raison des conditions de travail délétères des mineurs et des risques sanitaires importants qu’il engendrait. Le charbon Le charbon a ensuite été reconnu comme étant l’une des énergies les plus émettrices de dioxyde de carbone. En toute logique, la France a donc décidé de fermer ses mines de charbon. La dernière mine de notre pays a d’ailleurs cessé d’être exploitée en 2004 à Creutzwald, près de la frontière franco allemande. La fermeture de ces mines n’était toutefois qu’une première étape, puisque notre pays est encore doté de centrales à charbon. En 2020, quatre centrales à charbon étaient toujours ouvertes en France. Leur fermeture, annoncée en 2022, a été reportée à 2027 pour les deux dernières d’entre elles : les centrales de Saint Avold, en Moselle, et de Cordemais, en Loire Atlantique. En septembre 2023, le Président de la République Emmanuel Macron avait annoncé lors de la conclusion du Conseil de planification écologique l’ambition de décarboner notre économie et de réduire notre dépendance aux énergies fossiles.

d’une étape importante pour atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 et assurer notre souveraineté énergétique fondée sur le nucléaire et les énergies renouvelables. Conformément aux engagements pris par le Président de la République, il a donc été précisé à l’époque que les centrales à charbon de Saint Avold et Cordemais seraient converties au biogaz et à la biomasse d’ici à 2027.

converties à une autre source d’énergie primaire pour émettre moins de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure puissent être éligibles au futur mécanisme de capacité européen. Le texte présente selon moi de nombreux avantages, en matière de respect de nos engagements environnementaux, de renforcement de notre souveraineté énergétique ou encore d’emploi. Tout d’abord, il répond à une exigence essentielle, celle de respecter nos propres engagements environnementaux, en l’occurrence les accords de Paris, par lesquels la France s’est engagée à réduire significativement ses émissions de gaz à effet de serre.

réduire notre dépendance en la matière est décisif pour atteindre notre quête de souveraineté énergétique. En outre, faciliter la conversion d’une centrale à charbon présente des avantages non négligeables par rapport à la fermeture pure et simple d’un site. site. Bien évidemment, je me fais l’écho des arguments de l’auteur de la proposition de loi, qui soulignait en commission les conséquences sociales d’une reconversion. Environ 150 familles sont directement concernées, voire 500 familles si l’on prend en compte les emplois indirects. Dans des territoires déjà traumatisés par la désindustrialisation, lever les freins à la reconversion permettrait donc de préserver des centaines d’emplois sur les sites des anciennes centrales.

cinquante ans après l’apparition des premières centrales thermiques françaises et environ vingt ans après la fermeture de la dernière mine de charbon, nous discutons du devenir des deux dernières

à cette transition ; la garantie de notre autonomie énergétique et de nos approvisionnements en cas de pic de consommation, en cette période de hautes tensions internationales le respect des salariés et le maintien de leurs compétences rares d’énergéticiens. À ces conditions, nous ne pouvions que saluer la déclaration du Président de la République qui, le 23 septembre 2023, affirmait que Cordemais et Saint Avold allaient être reconverties

pour élaborer un projet de territoire commun, le négocier, le tester et convaincre. Dix ans pour soutenir la conversion de la plus grande centrale à charbon de France encore en activité autour du projet Ecocombust.

comme je l’ai rappelé ici même lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement du 16 octobre dernier. Une entreprise dont l’actionnaire unique est l’État ne peut dicter ainsi sa loi au politique et je ne ferai évidemment aucun commentaire sur l’actualité concernant la tête du groupe EDF… Par conséquent, nous ne pouvons que saluer la démarche transpartisane de notre collègue Khalifé Khalifé et des coauteurs de ce texte, ainsi que le travail

article est crucial pour conforter la transition énergétique et garantir la sécurité de l’approvisionnement de l’ensemble de nos territoires. Il impose à EDF de présenter un plan de conversion des centrales à charbon en lieux de production d’énergie à bas carbone d’ici à la fin

de notre souveraineté énergétique, de nos objectifs de transition et de la préservation de l’emploi dans nos territoires, mais aussi parce que l’on ne revient pas sur la parole présidentielle, nous serons particulièrement vigilants à la défense de cet article, lors de nos débats et tout au long du parcours parlementaire de cette proposition de loi. Je l’ai indiqué le 16 octobre dernier et je le répète aujourd’hui : la transition énergétique ne se fera pas contre les territoires et leurs habitants. Saint Avold et Cordemais doivent rester des lieux de production d’électricité. La parole

Il allait de soi que seule la conversion des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pouvait permettre une transition écologique socialement

Enfin, transpartisane et consensuelle, elle répondait aux attentes manifestées sur toutes les travées de la Haute Assemblée. La discussion générale de ce jour s’annonçait donc parfaitement sereine.

Surtout, cette décision, difficilement compréhensible, condamne la conversion de la centrale de Saint Avold et, avec elle, l’opportunité d’une véritable transition énergétique locale.

que le ministre de l’économie, répondant à ma collègue Catherine Belrhiti, qui l’interrogeait sur l’avenir du site de Saint Avold, a confirmé que la conversion de la centrale Émile Huchet en centrale à biomasse, trop complexe, serait remplacée par une conversion vers le gaz naturel ou le biogaz. Et le ministre d’expliquer que les « textes en vigueur ne permett[ai]ent pas d’opérer cette transformation à droit constant », ce qui impliquait la nécessité de légiférer.

parmi les nouvelles installations de production d’électricité et à s’assurer de l’éligibilité de celles ci au mécanisme de capacité de production d’électricité, prévu par le code de l’énergie.

Mes chers collègues, le maintien en activité d’une centrale permet de conserver le personnel sur place, de conforter le réseau des sous traitants et de ne pas engendrer de séisme socio économique sur le territoire. C’est un important facteur de stabilité, apprécié des élus, des décideurs et, surtout, de la population locale.

dans une filière énergétique d’avenir serait une erreur, non seulement économique, mais également écologique, dont nous serions tous comptables et que les générations futures ne nous pardonneraient pas.

son examen nous permet d’aborder la question de la sécurité de notre réseau électrique, de la gestion des pointes de consommation et de la conversion des centrales de production d’électricité à partir d’énergies fossiles, dans le cadre du mécanisme de capacité.

Oui, le changement climatique et les engagements de la France nous imposent de réduire, puis de supprimer, l’utilisation du charbon. Cela n’est pas remis en cause. Toutefois, nous avions imposé

; enfin, que les projets de conversion soient soutenus financièrement. Pour l’instant, il faut avouer que la gestion gouvernementale de ces fermetures laisse à désirer… Notre mix énergétique repose toujours sur une contradiction : l’augmentation nécessaire de la part des énergies renouvelables, par définition intermittentes, exige la présence de capacités pilotables, permettant de garantir l’équilibre du réseau.

En ce sens, les projets de conversion des deux dernières centrales à charbon, celles de Cordemais et de Saint Avold, relèvent non d’un fétichisme industriel, mais d’une nécessité dictée par les conditions objectives du réseau électrique.

chers collègues, sur le fait que le site de Saint Avold est détenu par une entreprise privée, propriété du milliardaire Kretinsky, dont on connaît les pratiques industrielles, à savoir toucher l’argent public puis liquider les outils de production.

Ecocombust est un projet de conversion industrielle, alliant préservation de l’emploi, développement de la filière et transition énergétique et écologique. C’est un projet vertueux, qui répond aux besoins de production électrique et aux enjeux climatiques. Il est donc inconcevable que l’État laisse

d’énergie. La pérennité de ces deux centrales répond avant tout à la nécessité de garder un filet de sécurité, même si, selon Réseau de transport d’électricité, en maintenant ou en convertissant ces centrales, « la couverture de leurs coûts d’exploitation [ne paraît] pas garantie ». Si ce n’était pas le cas, l’autre solution serait d’avoir recours à des importations d’électricité pour couvrir les pointes, à un prix bien plus élevé et avec un bilan carbone plus important. Enfin, au vu des débats de la commission des affaires économiques et de l’extension de l’accès au mécanisme de capacité à toutes les centrales thermiques, nous réitérons notre exigence d’un projet de loi consacré au futur de notre système électrique,… Absolument ! … en lieu et place du décret de programmation pluriannuel de l’énergie, qui prive le Parlement de sa compétence. La parole

l’histoire de la Moselle est intimement liée à ses industries et à ses mines. Le charbon y a façonné aussi durablement l’économie et le paysage industriel qu’il a coûté cher à ses habitants. Les friches minières, la pollution des nappes, les mouvements de terrain, les maladies respiratoires ou encore l’exposition à l’amiante constituent le lourd tribut payé par les mineurs et les Mosellans pour la reconstruction économique de la France. la France. Au siècle de l’écologie, nous ne pouvons pas simplement tourner la page de cette histoire comme celle d’un passé honteux et laisser dépérir ces régions industrielles sans proposer d’option de substitution viable et durable. Il nous faut résoudre cette équation complexe : en finir avec le charbon et les fossiles tout en garantissant la production d’électricité en période de tension et en préservant les emplois et le tissu industriel. Nous ne pouvons pas abandonner à leur sort les salariés, les ouvriers, les anciennes « gueules noires » et leurs ayants droit, car nous avons collectivement une dette envers eux. L’État a une responsabilité ; il a le devoir d’accompagner la transition de ces territoires, qui sont prêts à accueillir l’industrie verte de demain et la relocalisation de la production. Il ne s’agit pas pour autant de donner un blanc seing aux industriels, en se contentant d’engagements qui ne seraient pas respectés. La conversion de la centrale à charbon de Saint Avold est un enjeu social et écologique de taille et un pari risqué. Le projet de conversion en une centrale au gaz avec incorporation de 60 % de biométhane permettrait,, de réduire considérablement les émissions carbone du site. Tout dépendra de la provenance et du mode de production des 40 % restants, Nous veillerons particulièrement à ce que la centrale ne reste pas indéfiniment dans une phase transitoire, tournant uniquement aux énergies fossiles. L’effort pour la transition énergétique doit être partagé et il revient aussi à l’exploitant de tenir ses engagements. La réussite de ce projet de conversion est un enjeu économique et environnemental, mais surtout social. Des centaines d’emplois directs et indirects dépendent de ce site et sont aujourd’hui menacés. La confusion la plus totale quant à l’avenir de ces emplois est aggravée par les atermoiements sans fin des uns et des autres. L’État doit s’assurer que les salariés ne soient pas de nouveau victimes de mauvais choix industriels ou d’un manque d’anticipation. La conversion des dernières centrales à charbon correspond à un engagement présidentiel. Tout nouveau retard risquerait de compromettre définitivement la viabilité du projet et vouerait celui ci Nous voterons donc, de manière transpartisane, je l’espère, pour la suppression des dispositions susceptibles d’engendrer des délais supplémentaires. Nous soutiendrons également les amendements visant à éviter la mise en concurrence des centrales au fioul avec les centrales au charbon. La conversion de ces dernières, qui sont les plus polluantes, est plus complexe à mettre en œuvre et doit rester prioritaire. Tel est l’objet de cette proposition de loi. La décision de conversion des dernières centrales à charbon est un symbole important ; nous y adhérons, mais tout reste à faire et la bonne mise en œuvre de ce projet est cruciale si l’on ne veut pas discréditer notre ambition pour le climat et pour la justice sociale.

cet après midi pour évoquer un enjeu fondamental, qui engage à la fois notre souveraineté énergétique, la transition écologique de notre pays et l’avenir de centaines de salariés : la conversion de la centrale Émile Huchet de Saint Avold. Rappelons les faits. La loi Énergie Climat, promulguée en 2019, a acté la fermeture des centrales à charbon à l’horizon de 2022, marquant une avancée décisive dans notre lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, la crise énergétique provoquée par le conflit en Ukraine a bouleversé nos certitudes et a imposé des ajustements nécessaires.

Le 24 septembre 2023, le Président de la République a confirmé l’engagement du Gouvernement en faveur de la conversion des anciennes centrales à charbon. Cette annonce, qui s’inscrivait dans le cadre de la planification écologique, portait en elle une promesse, celle d’un avenir viable pour Saint Avold et ses salariés. Cette promesse s’est, hélas ! perdue derrière des lenteurs administratives. Alors que les salariés et les élus locaux attendaient un plan de transition concret, l’incertitude s’est installée, plongeant des centaines de familles dans l’angoisse et mettant en péril l’avenir du site.

qu’il tienne ses engagements. Saint Avold peut et doit devenir le symbole d’une transition énergétique réussie. Des projets concrets ont été présentés – production d’hydrogène, de gaz ou de biogaz – et les initiatives de l’exploitant du site témoignent d’une volonté d’adaptation et d’investissements massifs.

lever les blocages administratifs, garantir des procédures transparentes et offrir un cadre stable aux industriels et aux territoires concernés. Il est de notre responsabilité, en tant que législateurs, de faire en sorte que cette transition énergétique soit juste socialement et ne sacrifie ni les travailleurs ni la souveraineté énergétique de notre pays. En réponse à ma question d’actualité au Gouvernement du 12 février dernier, M. le ministre Lombard a confirmé le soutien du Gouvernement à la conversion de la centrale Émile Huchet au gaz et au biogaz. Cette déclaration a apporté un répit bienvenu aux salariés et a permis de prolonger les contrats pendants, en attendant le vote de cette proposition de loi. Il faut inscrire cette transition dans la durée, avec des décisions claires et irréversibles. En tant que législateurs, nous devons mettre fin à cette incertitude. Ce combat me semble important, ce texte ne doit pas être compromis. Il ne faudrait pas alourdir les procédures administratives et introduire des délais incompatibles avec la réalité économique et industrielle du projet.

qui avait promis la conversion des centrales à charbon. L’objectif de cette conversion est bien d’assurer une transition énergétique durable, non de favoriser des énergies fossiles encore plus polluantes. Mes chers collègues, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser ces modifications entraver un projet qui répond à des impératifs sociaux et d’urgence énergétique. Les pertes engendrées par les allongements de délai sont considérables – ils seraient d’environ 40 millions d’euros par an. Quel signal enverrions nous à l’ensemble des employés et à notre industrie si nous laissions les lourdeurs administratives mettre fin à un projet pourtant viable et essentiel ? Nous devons faire preuve de pragmatisme.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui nous donne l’occasion de consacrer la priorité numéro un dans le domaine de la transition énergétique poursuivre autant que possible la décarbonation ou la « défossilisation », voire, plus précisément encore, bien que nous soyons tenus à une certaine neutralité technologique, la « décharbonation » de notre mix énergétique. Au milieu d’un concert international parfois assourdissant, la France affiche un nombre ambitieux d’objectifs, tous plus difficiles à atteindre les uns que les autres, à des horizons dont on peine à déterminer s’ils procèdent d’une frénésie de marketing politicien ou d’une course ou d’une course à l’échalote avec nos pays voisins. Il est de bon ton, en effet, d’annoncer, à l’issue de conférences internationales, des conclusions fracassantes, marquées par le décalage entre les capacités réelles des États et les spéculations théoriques des négociateurs… Revenons à notre sujet. Chacun sait à quel point la France supporte largement la comparaison internationale en la matière, puisque les émissions natives de CO2 en France sont inférieures à six tonnes par habitant, contre quinze tonnes en Amérique du Nord ou en Chine. électrique, nous sommes même d’excellents élèves, puisque l’électricité produite sur notre sol est décarbonée à 95 %, principalement grâce à notre parc Vouloir « laver plus blanc que blanc » comporte le risque d’atteindre les confins de l’ubuesque, mais concédons que nos vertus réelles n’empêchent pas les efforts. Que reste t il donc à faire ? À mon sens, deux chantiers d’ampleurs très inégales. Idéalement, il reste d’abord à électrifier nos usages, c’est à dire à basculer des consommations énergétiques d’origine fossile vers la consommation de l’électricité vertueuse qui caractérise notre pays. Sur le papier, le schéma est assez simple, puisque c’est bien la part fossile du mix énergétique qui pèse encore lourdement dans notre bilan carbone. Dans la réalité, la chose n’est pas si aisée, parce que cela exige des investissements importants et que les industries manquent cruellement de visibilité tarifaire et politique. À l’évidence, l’instabilité récente dont souffre la tête du groupe EDF n’est pas de nature à les rassurer ; je ne suis pas marin, mais j’ai rarement vu un navire changer de capitaine au moment où il était indispensable de tenir la barre et de maintenir un cap.

Ces centrales ont joué un rôle capital au moment de la crise énergétique de 2022, en nous évitant un blackout redouté. À cet égard, je veux saluer les employés des sites, qui ont été rappelés en catastrophe

La solution la plus simple pour permettre cette transition consiste à installer des centrales au gaz. Le gain du point de vue des émissions de gaz à effet de serre serait très modeste, mais cela aurait l’avantage de la flexibilité.

serait source tant de vertus écologiques que de « pilotabilité ». En tout état de cause, le mécanisme de capacité doit pouvoir s’appliquer à toute forme de production inférieure au seuil de 550 grammes. La discussion

Merci

Cette disposition a suscité de vives inquiétudes en Moselle, car elle risque notamment de retarder de plus d’un an la conversion de la centrale de Saint Avold, compromettant ainsi la réussite du projet.

D’ailleurs, l’exposé des motifs de la présente proposition de loi indique déjà que le texte intervient à droit de l’environnement constant. En outre, il ressort de l’audition et de la contribution de la direction générale de l’énergie et du climat que l’autorisation environnementale n’est pas supprimée. Aussi, la commission demande le retrait des

Nous entendons les arguments du rapporteur selon lesquels l’article 3 ne constituerait en réalité qu’une coordination avec le droit existant et n’impliquerait pas de délai supplémentaire susceptible de freiner les projets de reconversion

Dans son audition et sa contribution, la direction générale de l’énergie et du climat a rappelé l’existence de négociations en cours avec la Commission européenne. De plus, elle a précisé qu’il serait préférable que la proposition de loi entre en vigueur en même temps que le nouveau mécanisme de capacité.

entrent en vigueur à une date fixée par décret et n’intervenant pas plus de six mois après l’approbation du dispositif par la Commission. Il serait en effet préférable que cette proposition de loi entre en vigueur à la même date que les évolutions du mécanisme de capacité, c’est à dire à la date prévue par décret, d’autant plus que cette proposition de loi renvoie à des articles qui ne seront

l’avis de la commission ? J’ai déjà mentionné la nécessité de conserver cette référence, qui garantit une bonne articulation de la proposition de loi avec la loi de finances pour 2025 et, au delà, avec la législation européenne sur les aides d’État.

Néanmoins, fixer l’obligation pour EDF de formuler un plan de conversion, c’est au fond lui imposer de prendre l’engagement suivant : cette conversion non seulement est possible, mais sera réalisée.

a annoncé sa volonté d’arrêter cette centrale d’ici à 2027, la conversion vers les pellets ou le gaz ayant été étudiée puis écartée pour des raisons technico économiques. L’amendement n° 33 du Gouvernement tend à préciser l’obligation

Vous êtes en train de dire qu’il faut une évaluation technique pour qu’il y ait un plan. Soit : vous enfoncez une porte ouverte ! On n’imagine pas un plan de conversion sans évaluation technique… Simplement, au lieu de

transition écologique tout le mal que je pensais de l’annonce qu’elle avait faite publiquement sans même rencontrer les organisations syndicales : elle était venue sur mon territoire pour annoncer la fermeture de la centrale

ont eu cette merveilleuse idée et que les polytechniciens qui sont à la tête d’EDF l’ont refusée que le groupe n’en a jamais voulu, malgré toutes les évaluations, et ce y compris – nous en avons la conviction – en faussant les chiffres

combien la désindustrialisation de la Moselle et la fermeture de ses mines, puis de ses hauts fourneaux, ont blessé – meurtri – ses habitants, toutes ces familles laissées sur le carreau.

Bien sûr, je pense à la centaine d’hommes et de femmes que j’ai pu rencontrer lors de mon passage à la centrale de Saint Avold. L’écologiste que je suis sait que le gaz produit inefficacement de l’électricité.

modifié, l’ensemble de la proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement. Mes chers

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat examine aujourd’hui la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale visant à renforcer les conditions d’accès à la nationalité française française à Mayotte. Nul n’ignore ici la situation exceptionnelle que connaît ce territoire français, le plus jeune jeune de nos départements, confronté à des flux migratoires d’une intensité inégalée, à des tensions sociales croissantes et à une pression démographique qui met à rude épreuve l’ensemble de ses services publics, son tissu social et son développement économique, en un mot, la République.

et la possibilité actuelle d’acquérir la nationalité française par simple effet du droit du sol ont transformé cette île en porte d’entrée de l’immigration irrégulière vers la République. Les chiffres parlent d’eux mêmes : près d’un habitant sur deux à Mayotte est de nationalité étrangère. Chaque année, des milliers de femmes enceintes prennent tous les risques pour accoucher sur le territoire, animées

mesure est essentielle pour prévenir les reconnaissances frauduleuses de paternité, devenues trop nombreuses. Il revient au Sénat de rétablir un équilibre : l’accès à la nationalité française ne saurait découler d’une simple présence de fait,

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 6 septembre 2018, a reconnu la spécificité de Mayotte et la légitimité d’une adaptation du droit sur le sol mahorais. Il nous a donné un cadre : les mesures doivent être limitées, adaptées et proportionnées.

Mesdames, messieurs les sénateurs, votre Haute Assemblée a toujours su porter un regard lucide et exigeant sur les équilibres constitutifs de notre République. Elle a toujours été attentive à l’adaptation du droit sur tous les territoires,

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, Mayotte est confrontée, depuis plusieurs décennies, à une intense pression migratoire. Parmi les 320 000 habitants qui peuplent cette île, on compte ainsi 50 % de ressortissants étrangers, dont la moitié serait en situation irrégulière.

qui est le plus important, en provenance des Comores, donne lieu à l’arrivée d’environ 20 000 migrants en situation irrégulière chaque année. Cette immigration, qualifiée par le préfet de Mayotte

de l’île ne doit pas être sous estimée. Mayotte fait partie intégrante de l’archipel des Comores et est située à seulement 70 kilomètres

En 1974, lorsque Valéry Giscard d’Estaing décide de consulter les Comores sur leur indépendance, trois îles comoriennes affirment une volonté d’indépendance, à plus de 99 alors que le résultat sur l’île de Mayotte est inverse et beaucoup plus nuancé, 63 % de ses habitants souhaitant rester dans la République. Ce résultat est essentiel à la compréhension du problème actuel. En effet, la majorité des Mahorais ont conservé des liens familiaux et culturels avec les Comores, ce qui donne lieu à de nombreux échanges et flux migratoires.

en place, avec un groupe d’élèves scolarisés le matin, et un autre l’après midi. Les effets sont également visibles dans le domaine de la santé, l’offre de soins ne pouvant absorber continuellement une croissance démographique exponentielle.

D’après une estimation des services des douanes et de l’Institut d’émission des départements d’outre mer (Iedom), 100 millions d’euros circuleraient annuellement entre Mayotte et Anjouan, soit 100 millions d’euros qui manquent cruellement à la demande intérieure. Enfin, l’immigration à Mayotte pose des difficultés sanitaires. On observe par exemple la résurgence de maladies qui avaient disparu, en raison d’une absence de vaccination chez les enfants en situation irrégulière.

et déjà se féliciter que le nombre d’acquisitions de la nationalité française au titre du droit du sol ait diminué assez significativement depuis son entrée en vigueur, passant de près de 3 000 en 2018 à 800 en 2022.

lieu, la commission a supprimé l’obligation pour le parent de présenter un passeport biométrique à l’officier d’état civil à la naissance de l’enfant, pour permettre l’apposition sur l’acte d’une mention relative à la durée de séjour régulier dudit parent en France. Cette mention est censée faciliter par la suite les démarches d’acquisition de la nationalité française par le biais du droit du sol.

Seule une réponse globale pourrait réduire significativement les flux migratoires à destination de l’archipel. Cette réponse globale pourrait par la mise en place effective du « rideau de fer » imaginé dès février 2024 par l’ancien ministre de l’intérieur un durcissement des conditions d’obtention des titres de séjour ; ou encore la conduite d’une politique de coopération avec les Comores pour les accompagner dans un développement intelligent

qui dissuadera sans aucun doute certains candidats à l’immigration, pour qui l’accès éventuel à la nationalité constitue un réel facteur d’attractivité. C’est pourquoi, mes chers collègues, au bénéfice de ces observations, je vous invite à adopter la proposition de loi, ainsi modifiée. Nous passons

Avec une loi visant à restreindre l’accès à la nationalité française, vous ne répondrez en rien aux besoins de la population mahoraise. Dire aux Mahorais, qui doivent faire face à des difficultés d’accès à l’eau, à la santé, à l’éducation et à tous les services publics, qu’une réforme du droit du sol améliorera leur quotidien

de citer l’article 73 de la Constitution de 1958 : « Dans les départements et les régions d’outre mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités. Mayotte fait partie de la République française. À ce titre, les principes républicains et constitutionnels doivent s’y appliquer, comme dans tous les territoires français, dans l’Hexagone comme en outre mer.

sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. » Édicter des dispositions discriminatoires et spécifiques au seul territoire mahorais, c’est, en substance, renouer avec une approche coloniale de la nationalité française. Nous refusons de revenir à un droit de la nationalité discriminatoire en outre mer ! Je tiens à insister sur le caractère disproportionné et inefficace de ce texte. Nous n’avons pas besoin de prévoir un nouveau durcissement de la loi Asile et Immigration de 2018. Celle ci dispose qu’un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne peut acquérir la nationalité française que si, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins résidait en France de manière régulière depuis trois mois.

ailleurs, cette loi de 2018 n’a jamais eu le moindre effet sur les migrations. Le ministère de l’intérieur assure que le nombre d’acquisitions de la nationalité française a été divisé par trois, passant de 2 900 en 2018 à 860 en 2022. Or les flux migratoires, eux, se sont intensifiés depuis. En réalité, l’accès à la nationalité est loin d’être la principale cause des migrations. Par le biais de cette proposition de loi, vous souhaitez dissuader les mères étrangères de venir donner vie à Mayotte. la réalité, c’est qu’aucun étranger ne consultera les dispositions de ce texte avant d’immigrer à Mayotte ! Ce qui motive le départ pour cette île, c’est l’espoir d’une vie meilleure, le rêve de voir ses enfants aller à l’école, la peur, aussi, de mourir en accouchant si on le fait

en situation irrégulière à Mayotte ; vous ne ferez que créer de la clandestinité ! Et créer de la clandestinité, c’est augmenter la précarité. Je rappelle que les résidents étrangers sont, pour la moitié d’entre eux, en situation régulière, et vivent à Mayotte depuis longtemps. Ils occupent des emplois formels. Ils assument des tâches difficiles et essentielles, dans les champs ou sur des chantiers. Ceux à qui l’on refuse des papiers doivent occuper des emplois informels, dans des conditions de travail indignes et illégales. qui m’est donnée de m’exprimer pour dénoncer une irrégularité créée artificiellement par le manque d’accessibilité des services préfectoraux. Depuis deux ans, la préfecture de Mayotte ouvre rarement ses portes. s’ajoute à la dématérialisation des demandes de titres et à l’obligation de prendre les rendez vous en ligne. Entraver une personne dans sa démarche de régularisation revient à aggraver sa précarité, à l’exclure de la société et à la plonger dans la clandestinité. proposition de loi contre productive. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2018, le nombre d’acquisitions de la nationalité a baissé. Je vous le demande, en quoi cela a t il amélioré la situation de l’île ?

que l’immigration comorienne menace la culture mahoraise, c’est faire fi de l’histoire du peuple comorien. Comoriens et Mahorais partagent une même culture, une même langue, une même religion, une même organisation matrilinéaire.

unique dans le pays. Nous considérons que, sans être l’unique facteur d’une situation éminemment complexe, les conditions d’accès à la nationalité française par le mécanisme du droit du sol ont contribué à renforcer l’attractivité de ce territoire comme destination de ces flux.

Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 septembre 2018, portant précisément sur le dispositif en vigueur, ce dernier ne méconnaît ni le principe d’égalité devant la loi ni les exigences découlant de l’article 1 de la Constitution.

à l’identité française, mais pour protéger l’identité kanake. Il s’agissait d’un processus de décolonisation et de construction de la citoyenneté calédonienne. Cela n’a rien à voir avec la situation du territoire de Mayotte, qui a choisi de rester français et d’entrer

un lien entre le droit de la nationalité et l’immigration, a durci les règles d’accès à la nationalité française à Mayotte. Elle prévoit ainsi, par dérogation au droit commun, qu’un enfant né à Mayotte ne peut obtenir la nationalité française

au contraire. En 2022, le nombre de nouveau nés ayant une mère étrangère était même supérieur de 14 % par rapport à 2018. En 2023, le nombre d’étrangers interpellés en mer a augmenté de 128 % par rapport à 2020. Cela

Aucune réforme législative ou réglementaire relative à la nationalité ne pourra changer cela ! C’est d’ailleurs ce qu’indique, en creux, le rapport de la commission des lois du Sénat sur ce texte : « Si cette réforme – celle de 2018 – a permis de diminuer le nombre d’acquisitions de la nationalité française au titre du “droit du sol”

« un enfant né en France est Français. C’est notre histoire. C’est notre tradition. C’est comme ça que la France est devenue un grand pays. » Ces mots sont de… Nicolas Sarkozy. La seconde raison,

allonger le maintien en rétention de personnes condamnées ; créer une condition de durée de résidence pour obtenir des prestations sociales ; complexifier l’exercice du droit de vote pour les personnes emprisonnées ; interdire le mariage lorsque l’un des futurs époux est en situation irrégulière sur le territoire français ; interdire

pas parce que vos connaissances en droit constitutionnel seraient défaillantes, mais parce qu’au fond la Constitution et ses principes vous dérangent.

Or la Constitution est un rempart contre les discriminations, contre le racisme et contre l’arbitraire. Dans votre fuite en avant décomplexée vers la remise en cause de ce qui a fait ce dont la France peut être la plus fière, épargnez, s’il vous plaît, les Mahoraises et les Mahorais ! Mayotte ne mérite pas d’être ainsi

personne n’a rien à gagner à voir s’effriter l’État de droit et les valeurs de la République. Mayotte a besoin que la République lui soit utile, et non d’être utilisée pour détricoter la République ! La parole

L’archipel mahorais devra en effet faire l’objet de mesures législatives spécifiques et ambitieuses. Le moment venu, nous participerons bien sûr pleinement à leur discussion.

décider de son avenir.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cette proposition de loi qui nous vient de l’Assemblée nationale a fait couler beaucoup d’encre et de salive

Objectivement, les résultats de la lutte contre l’immigration démontrent l’échec patent de cette politique publique à Mayotte. Pour illustrer mon propos,

: la suppression des cartes de séjour territorialisées pour les étrangers en situation régulière. Selon les chiffres officiels, près de 90 000 étrangers en situation régulière sont assignés à résidence à Mayotte.

aurez prochainement à vous prononcer sur cette mesure, qui aura des effets très concrets sur la vie quotidienne des Mahorais et sera bénéfique pour les finances publiques. La

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame la présidente de la commission des lois, mes chers collègues, Mayotte souffre, et sa souffrance ne date pas du passage dévastateur du cyclone Chido. Elle dure depuis des années, nourrie par une immigration massive, incontrôlée et destructrice de la paix publique comme de la prospérité. Malgré les visites officielles, malgré les opérations Wuambushu et malgré les promesses répétées, les gouvernements successifs ont failli. Par mépris pour un territoire jugé lointain ou par idéologie, ils ont échoué à protéger Mayotte et ses habitants. Ce département, le plus pauvre de France, est submergé par une immigration anarchique, abandonné par ceux qui, à Paris, détiennent les moyens d’agir. L’insécurité y est insoutenable, les services publics y sont exsangues et les Mahorais eux mêmes se sentent étrangers sur leur propre terre. Qui peut tolérer que des Français vivent ainsi dans la peur des vagues d’immigration clandestine ? Chaque jour, de nouveaux migrants franchissent la frontière maritime depuis les Comores. La réalité, mes chers collègues, c’est que Mayotte est un territoire au bord de l’explosion. Près de la moitié de sa population est étrangère. Chaque année, des milliers d’enfants y naissent de parents en situation irrégulière, profitant du droit du sol pour obtenir la nationalité française. Les conséquences sont connues : un hôpital saturé, un système social débordé et une criminalité endémique, menaçant le quotidien des habitants. Ce constat, Marine Le Pen l’a fait depuis longtemps. Ah ! En 2018 déjà, elle lançait l’alerte en déposant une proposition de loi spécifiquement dédiée à ce sujet. Elle a écouté la détresse des Mahorais et leur a adressé un message clair : nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous trahirons pas.

Mayotte est aujourd’hui le présage de ce qui menace la France si nous ne réagissons pas. La situation y est hors de contrôle, et elle préfigure ce qui nous attend si nous laissons l’immigration de masse détruire notre cohésion nationale.

elle est à la fois sociale, sanitaire, sécuritaire et institutionnelle et met aujourd’hui en péril notre pacte républicain. Les Mahorais n’en peuvent plus. Ils ont le droit de vivre dignement, en sécurité, et dans le respect des principes qui fondent notre République. Ils doivent bénéficier, au même titre que tout citoyen français, de la justice et de la sécurité. Or l’immigration irrégulière massive sature les infrastructures La violence, croissante, et l’économie informelle gangrènent la société mahoraise. Accès à l’eau, à l’électricité, à l’éducation ou encore aux soins : rien n’est garanti, tout est devenu l’objet de luttes quotidiennes. Avec plus de 10 000 naissances chaque année, Mayotte occupe le deuxième rang des départements français en matière de natalité. Les trois quarts des mères y sont toutefois de nationalité étrangère. Quant au système hospitalier, il y est à bout de souffle. L’hôpital de Mamoudzou croule sous les urgences et les pompiers interviennent pour des centaines d’accouchements hors maternité. n’est plus tenable. Face à cette réalité, le droit du sol, tel qu’il s’applique aujourd’hui à Mayotte, ne fonctionne plus ; et pour cause, il a été détourné. Alors que la population vit un enfer, les passeurs, eux, se frottent les mains. Les reconnaissances de paternité frauduleuses sont légion ; on dénombre même parfois plusieurs dizaines de reconnaissances par père.

Il nous faudra également renforcer les moyens de lutte contre l’immigration clandestine en exigeant une coopération accrue des Comores. Les infrastructures, notamment le réseau de transport, devront être modernisées, comme dans de nombreux autres territoires ultramarins –, il faudra réinterroger le modèle économique local afin de créer de l’emploi et de sortir de l’économie informelle.

l’insécurité, l’insalubrité, la dégradation de l’environnement et des ressources, l’aggravation des problèmes sanitaires ou encore la saturation des services publics. Les femmes, inquiètes pour elles mêmes comme pour leurs enfants, sont souvent en première ligne dans ce combat. Il aura fallu les images terribles prises après le passage du cyclone Chido pour que les Français de métropole voient concrètement l’état de Mayotte, ses collines déforestées où des milliers de familles s’entassent dans des baraquements insalubres et illégaux. L’accroissement incontrôlé de la population, couplé à l’accélération de bouleversements climatiques suscitant eux mêmes des flux migratoires, représente un risque majeur pour l’avenir de Mayotte. Au delà de l’augmentation des flux, on constate la diversification de l’origine des migrants qui rejoignent ou tentent de rejoindre Mayotte.

En 2018, le législateur a ajouté une condition spécifique à Mayotte pour l’acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers. Il a exigé qu’au moment de la naissance l’un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois mois. Ces dispositions figurent à l’article 2 493 du code civil. Le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution, en reconnaissant qu’il existe à Mayotte Mayotte « une forte proportion de personnes de nationalité étrangère, dont beaucoup en situation irrégulière, ainsi qu’un nombre élevé et croissant d’enfants nés de parents étrangers ».

Enfin, la commission a supprimé l’obligation de présentation d’un passeport biométrique à l’officier d’état civil par le parent étranger, car tous les pays n’en disposent pas. Il me semble que ces mesures équilibrées devraient contribuer à réduire la pression à Mayotte. L’autre sujet que je souhaite évoquer est d’ordre géopolitique. Il est lié aux bouleversements de l’ordre mondial en cours. depuis plusieurs années, certains de nos compétiteurs et leurs vassaux ont développé des stratégies hybrides pour contester notre présence dans certaines espaces géographiques. Ces espaces, d’un intérêt stratégique ou économique réel, sont de plus en plus convoités. C’est le cas de nos outre mer et de leurs zones économiques exclusives (ZEE), que la France, avec ses moyens modestes, peine à surveiller et à protéger. La présence française dans le sud de l’océan Indien et le canal du Mozambique est ainsi une cible clairement identifiée. En s’appuyant sur un narratif anticolonial, sur de la propagande et de la désinformation, ces discours façonnent un environnement cognitif hostile à la France. Cela fonctionne : regardons ce qui se passe actuellement dans certaines zones de l’Afrique francophone, voire en Nouvelle Calédonie. Chacun a aussi pu observer comment certaines puissances instrumentalisent les flux de migrants vers l’Europe, pour fragmenter les sociétés et créer une situation de chaos. Cette stratégie indirecte, je vous l’assure, n’est pas une vue de l’esprit elle figure clairement dans la doctrine d’action de plusieurs pays. Dans le contexte dégradé de Mayotte, l’immixtion de rivaux stratégiques et leur rapprochement intéressé avec des États voisins ont de quoi inquiéter. Dans leur propre intérêt, ces compétiteurs soutiennent la « restitution » de Mayotte aux Comores, ainsi que celle des îles Éparses à Madagascar. Pour eux, tous les moyens de déstabilisation sont bons, qu’ils soient informationnels, de droit

je m’exprime aujourd’hui en tant que représentante de Mayotte, un territoire confronté à une pression migratoire et à un traitement de la question migratoire sans équivalent dans notre République.

fausse les données démographiques et masque les besoins réels de la population mahoraise. Cette situation compromet également l’accès légitime des Mahorais et des Mahoraises aux infrastructures publiques essentielles.

Par ailleurs, la suppression de l’exigence de résidence pour les deux parents, une décision qui vise à éviter toute discrimination à l’égard des familles monoparentales, soulève des inquiétudes. l’une des raisons pour lesquelles le rapporteur a souhaité rétropédaler est pourtant déjà très prégnante sur le terrain. Ainsi, le recours à un père de nationalité française le temps d’un instant,

Ne vous méprenez pas, les reconnaissances frauduleuses de paternité sont déjà largement répandues dans les circonstances actuelles. Le retour à la rédaction initiale du code civil nous laisse penser que la réforme annoncée a été délaissée au profit d’un simple agencement des règles existantes. L’ambition s’est égarée en

Aussi, j’appelle le Gouvernement à se saisir de cette demande de réforme dans le cadre du futur projet de loi pour Mayotte en cours de préparation. sans une réponse de fond à cette problématique, tous les efforts des uns et des autres seront vains. Pour faire face à la saturation à laquelle Mayotte est confrontée et dans l’attente d’un projet de loi téméraire, cette proposition de loi constitue, par défaut,

par des moyens encore accrus sur le terrain pour endiguer les flux migratoires et, enfin, répondre à la demande initiale des Mahorais, qui luttent pour se réapproprier leurs terres et leurs droits.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, « la France est une République indivisible ». Une phrase, six mots d’une concision et d’une précision exemplaires, inscrits à l’article 1 de notre Constitution.

Donc, lorsque le Président de la République affirme que « Mayotte est la première maternité de France, avec des femmes qui viennent y accoucher pour faire de petits Français », il se trompe. Il faut mettre fin à ce fantasme auquel on veut faire croire, à tort, nos concitoyens : ce n’est pas parce que l’on naît à Mayotte que l’on devient Français. ne s’agit pas d’une vue de l’esprit, mais d’une réalité juridique. Troisième fait à établir : Mayotte doit faire face à un incommensurable problème d’immigration. Cette immigration, comme le rapporteur nous l’a expliqué, vient des pays voisins, et principalement des Comores, dont Mayotte faisait partie jusqu’au référendum de 1974. La moitié des enfants nés à Mayotte sont issus de couples mixtes, comprenant

La question qui se pose, la seule question intéressante d’ailleurs si l’on cherche des solutions, est la suivante : pourquoi les migrants vont ils à Mayotte ? Ils n’y vont certainement pas pour obtenir un passeport : il a été rappelé que ce n’était pas si simple. Ils y vont, car les liens familiaux y sont déjà intenses, car la culture, y compris la religion, est commune

Nous avons donc créé, en plein milieu de l’océan Indien, une frontière entre le Nord et le Sud. Mayotte est huit fois plus riche que les Comores. Cet écart de développement est comparable à celui qui existe entre les États Unis et le Mexique.

Pour autant, nous ne pensons pas que c’est en modifiant une seconde fois notre droit du sol spécifiquement pour Mayotte, sans même avoir pu évaluer l’impact du changement décidé en 2018, que nous arriverons à stopper l’immigration illégale. D’ailleurs, les chiffres indicatifs dont nous disposons ont plutôt tendance à montrer que cela n’a rien changé en termes de flux migratoires. évidemment, la situation actuelle est insupportable pour les Mahorais. Mais, pour y remédier, notre droit n’y pourra rien. Alors, plutôt que de ronger encore un peu plus ce principe structurant de notre peut être pourrions nous engager une véritable politique publique visant à s’attaquer aux réelles causes de l’immigration illégale et massive : la pauvreté aux Comores. Cette politique existe. Elle a même un nom, souvent décrié aujourd’hui, alors que nous avons là un exemple patent de son utilité : l’aide publique au développement. Parce que la réponse à apporter à Mayotte n’est, malheureusement, pas juridique, et parce que mon groupe est radicalement républicain, nous refuserons de voter cette proposition de loi ! La parole

Deux objectifs majeurs ont guidé la réflexion de nos deux collègues : s’interroger sur la capacité de l’État à assurer pleinement ses missions fondamentales et engager des politiques publiques permettant de répondre efficacement aux réalités des territoires et, avant tout, aux besoins et aux attentes des habitants. Or lutter contre l’immigration clandestine est une demande constante exprimée par les Mahorais. Pour y répondre, la recommandation n° 22 dudit rapport vise à réexaminer le mode d’acquisition de la nationalité française par les enfants nés à Mayotte de parents étrangers, en envisageant de revoir la durée exigée de résidence régulière et ininterrompue sur place des deux parents, avant la naissance.

Il ne suffit ainsi pas de naître en France pour être Français d’origine, autrement dit Français de plein droit à la naissance. La nationalité est attribuée en principe, parce qu’au moins l’un des parents est Français. Le droit du sol ne joue qu’un rôle

Comme l’ont écrit plusieurs auteurs, la mesure proposée pour Mayotte pourrait très bien s’appliquer à d’autres parties du territoire national si des circonstances particulières le justifiaient, et ce en vertu de l’article 73 de la Constitution.

effet, puisque ce type de document n’est délivré que par un nombre limité d’États, l’application de cette mesure aurait pu être source de discriminations selon le pays d’origine.

Le véritable enjeu serait l’accession à la nationalité française des enfants nés sur l’île et y ayant passé dix huit années. Pourtant, aucun chiffre, aucune analyse ne permet de démontrer que les conditions d’accès à la nationalité à Mayotte

qui enferment et condamnent encore davantage ses habitants. C’est le cas des titres de séjour délivrés à Mayotte, qui ne permettent pas de circuler librement sur l’ensemble du territoire français et dans l’espace Schengen. La population de Mayotte est abandonnée par notre État et discriminée par nos lois. Et pourtant, Mayotte s’inscrit dans une géographie et dans une histoire trop souvent ignorées pour servir des intérêts électoraux. Ainsi, l’archipel des Comores est composé des îles d’Anjouan, de la Grande Comore, de Mohéli et de Mayotte. de Mayotte. À l’amorce du processus d’indépendance des Comores en 1974, l’archipel est encore considéré dans son entièreté, et c’est le peuple comorien uni qui est appelé à se prononcer lors du référendum. Valéry Giscard d’Estaing, alors Président de la République, le rappelait en ces termes : « les Comores sont une unité, ont toujours été une unité. […] Nous n’avons pas, à l’occasion de l’indépendance d’un territoire, à proposer de briser l’unité de ce qui a toujours été l’unique archipel » des Comores. Cependant, après le référendum, le gouvernement français adopta une attitude opposée, interprétant les résultats à son avantage et s’assurant de garder une position stratégique dans le canal du Mozambique, au détriment de l’unité du peuple. dans l’ensemble de l’archipel, plus de 95 % du peuple comorien s’était prononcé en faveur de l’indépendance. Mais, en son sein, les habitants de l’île de Mayotte avaient voté à 65 % contre l’indépendance. L’État français a alors divisé l’archipel et le peuple comoriens. Aujourd’hui cette histoire résonne. Il y a eu deux votes

d’abord, parce qu’elle détourne l’attention d’une catastrophe humanitaire, sociale et écologique sans précédent à Mayotte. Elle est indécente ensuite, parce qu’elle instrumentalise la détresse des Mahoraises et des Mahorais au profit, j’ose le dire, d’une stratégie électorale dangereuse. indécente enfin, parce que Mayotte souffre. Et face à cette souffrance, quelle est votre réponse ? Durcir encore l’accès à la nationalité ? Restreindre encore un peu plus le droit du sol ? Ajouter de nouvelles contraintes aux enfants nés à Mayotte ? Quelle indécence ! Mayotte est un département de la République que vous traitez comme une exception permanente, comme le territoire de toutes les régressions. Depuis 2018, les conditions d’accès à la nationalité française y ont déjà été réduites par la loi Collomb. Cette dérogation territoriale impose déjà des critères plus stricts aux enfants nés à Mayotte.

de priver de nombreux jeunes d’une nationalité à laquelle ils avaient droit, de fabriquer des « invisibles », de créer une citoyenneté de seconde zone.

d’une crise écologique ensuite, avec des ressources en eau épuisées, une gestion des déchets chaotique et un territoire asphyxié par l’absence d’infrastructures adaptées.

détruisant des milliers de foyers, arrachant les toits, inondant les terres, laissant un paysage de désolation derrière lui. Face à cette situation d’urgence absolue, l’action de l’État

; reconstruire, pour donner un avenir durable à Mayotte, en investissant massivement dans les infrastructures et en mettant fin aux politiques d’exception, qui condamnent l’île à l’abandon. Ce texte ne répond en rien aux défis auxquels Mayotte

une faiblesse. C’est une conception de la nation, qui repose sur l’inclusion et l’intégration. Vous voulez faire croire que l’immigration est le problème, alors que le véritable problème de Mayotte est son abandon par l’État. Depuis plusieurs mois, votre majorité multiplie les attaques contre les étrangers et contre les principes républicains. Hier, vous avez voulu interdire le port du voile dans le sport, et aujourd’hui, vous vous en prenez au droit du sol. À force de relayer les obsessions de l’extrême droite, vous lui préparez le terrain, avec ses thèmes, vous normalisez son discours. Alors, nous allons nous battre pour nos valeurs républicaines : nous allons nous battre dans cet hémicycle ; nous allons nous battre dans la rue nous allons nous battre partout, parce que nous refusons cette musique nauséabonde de l’exclusion et du rejet de l’autre ! La France a besoin de solidarité, pas de discrimination

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Républicains, soutenu par le Gouvernement, nous propose aujourd’hui de revenir sur le droit du sol à Mayotte, poursuivant ainsi sa confusion progressive, voire sa fusion, avec l’extrême droite. passage du cyclone Chido, qui a dévasté Mayotte, et face aux terribles problèmes qui touchent le territoire – manque d’investissements chronique fragilisant les services publics, déficit criant de logements décents, absence d’accès à l’eau potable –, certains ici estiment avoir trouvé la solution.

Depuis 1515, le droit du sol permet à l’enfant d’un étranger né et résidant en France de devenir Français. En 1889, ce principe est devenu un fondement de la République. Patrick Weil a dit Le droit du sol républicain, progressif et conditionnel, est tellement au fondement de notre identité nationale que même le régime de Vichy l’a maintenu dans le projet de réforme de la nationalité qu’il avait préparé. Contrairement à ce que certains prétendent dans notre hémicycle, le simple fait de naître sur le territoire français ne confère pas la nationalité française. Il n’y a aucune automaticité pour les enfants qui naissent sur le territoire mahorais. C’est la double condition cumulative de la naissance couplée à la résidence en France au moment de la demande et pendant au moins cinq années durant l’adolescence, qui permet d’acquérir la nationalité française. Vous nous Vous nous proposez donc de violer l’indivisibilité de notre République, après l’avoir fait une première fois en 2018 la loi Asile et Immigration.

En dépit de nombreuses demandes formulées par des parlementaires, il n’existe aucune évaluation du régime dérogatoire mis en place en 2018 qui permette de mesurer l’effet escompté sur l’immigration irrégulière. Pire, si le nombre des acquisitions de la nationalité française à Mayotte à la majorité a été divisé par trois, celui des étrangers en situation régulière a été multiplié par dix. Quant au nombre de naissances sur l’île, il n’a cessé d’augmenter, avec une hausse de 47 % entre 2014 et 2022. Comment osez vous sérieusement prétendre qu’il existe une corrélation entre le droit de la nationalité et la lutte contre l’immigration régulière ? J’ai souvent l’impression, chers collègues de droite, que votre aveuglement vous empêche de vous mettre à la place de ces hommes et de ces femmes qui fuient les Comores et d’autres pays de la région et de vous poser

préférez plutôt imaginer ces personnes en train de peser le pour et le contre d’une traversée où elles risquent leur vie en se demandant si leurs futurs enfants pourront bénéficier de la nationalité française… Quelle déconnexion et quel cynisme ! Je le dis à ce gouvernement et à certains qui se croient encore de gauche sur une partie des travées de notre Avec cette réforme, vous violez une fois de plus notre Constitution. L’atteinte manifeste et disproportionnée de cette proposition de loi au droit du sol n’est ni justifiée ni adaptée. Il n’a jamais été démontré, depuis 2018, que la réforme du droit du sol avait endigué les flux migratoires. Au contraire, elle n’a fait qu’accroître la grande précarité de nombreuses familles et de jeunes privés d’accès à la nationalité française

et nous comprenons bien pourquoi : ce texte est d’abord un tract politique ! Il n’a pas pour objet d’apporter une réponse juridique solide aux difficultés que rencontrent Mayotte et les Mahorais. Avant d’envisager toute modification du droit de la nationalité à Mayotte, la priorité aurait été d’évaluer la loi de 2018 et la restriction du droit du sol qui s’applique

Ce qui paraît évident pour tout le monde ne l’est donc ni pour la commission des lois, qui se retranche derrière le rejet habituel des demandes de rapport, ni pour le Gouvernement, qui, depuis cinq ans, fait obstruction à toute évaluation de la loi de 2018. Je relève d’ailleurs que le groupe RDPI lui même, qui défendait le principe d’une évaluation en 2024,

pendant les trois mois précédant la naissance de l’enfant. Ce document devra analyser les conséquences de la loi sur les droits des enfants, les flux migratoires et l’évolution du nombre de titres de séjour délivrés à Mayotte. Le texte que nous étudions aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des mesures de 2018 renforce, sans que nous les ayons évaluées. Modifier un principe aussi fondamental que le droit du sol nécessite pourtant de juger les impacts d’une telle réforme. Les premiers résultats dont nous disposons sont les chiffres du ministère du ministère de l’intérieur et des professionnels sur le terrain. Ils ne démontrent pas que les durcissements législatifs précédents ont répondu à l’objectif des pouvoirs publics d’endiguer les flux migratoires. Nous l’avons dit, ce texte nous semble par ailleurs comporter des menaces sérieuses pour les droits des enfants.

on ne peut pas procéder à des adaptations de la loi qui n’ont aucun lien avec les difficultés du territoire. Or c’est exactement ce qui est proposé dans ce texte. Nous n’allons pas résoudre les difficultés migratoires à Mayotte en remettant en cause le droit de la nationalité.

un traitement différencié et injustifié, fondé sur l’origine. Une telle disposition est proprement discriminatoire. Elle va à l’encontre du principe d’égalité entre tous, qui est proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

retrouvent piégés à Mayotte et ont pour seul sort les bidonvilles, la peur, la faim et la haine. Il y a moins d’une semaine, nous votions à l’unanimité une résolution visant à mettre fin au sans abrisme des enfants.

à défaut d’appliquer le principe de solidarité qui prévaut pourtant entre tous les territoires européens.